La séance est reprise. La parole est à M. Bernard Delcros, pour une mise au point au sujet d'un vote.

Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au et figurera dans l'analyse politique du scrutin. L'ordre du jour appelle une déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, portant sur le projet de programme de stabilité pour 2018-2022, en application de l'article 50-1 de la Constitution.

! En matière de croissance, nous pouvons et nous devons faire encore mieux. Notre niveau de chômage structurel reste supérieur à la moyenne des pays de l'OCDE. Notre déficit commercial se creuse depuis 2001 sous l'effet des pertes de compétitivité.

La voie consistant à augmenter systématiquement la dépense publique, comme certains le proposent, a donc déjà été explorée : c'est une impasse ! Quant à nous, nous voulons tenter autre chose, pour éviter d'avoir toujours plus de dépenses publiques,

une démarche de réduction de la dépense publique et une démarche de transformation structurelle de notre économie. C'est en avançant sur ces deux jambes que nous pourrons rétablir la prospérité en France. Il ne s'agit pas de tailler dans les dépenses publiques pour tailler dans les dépenses publiques, ou de faire des réformes économiques pour faire des réformes économiques. Il s'agit, à la fois, de rétablir nos finances publiques et de permettre à notre appareil de production de se moderniser, d'innover, de créer des emplois,

besoin de capitaux ; il faut en mettre à leur disposition. Nous avons aussi réformé le marché du travail. Nous allons poursuivre ces transformations au travers du projet de loi sur la croissance et la transformation des entreprises, qui vise à rendre notre tissu productif

de rester une nation technologiquement souveraine. Je souhaite que, demain, nos véhicules autonomes soient pilotés par des systèmes européens, et non chinois ou américains.

Nous n'accomplissons pas ces transformations économiques pour que ceux qui réussissent déjà réussissent toujours mieux ; nous les faisons pour que chaque Français, d'où qu'il vienne,

fait des bénéfices. C'est une question de justice, c'est une question d'équité ! L'intéressement et la participation, nous n'en parlons pas, nous les faisons.

Le quatrième aspect de ces réformes structurelles, c'est la transformation de l'État. En effet, il va de soi, pour nous, que la transformation économique du pays passe par une redéfinition des rôles respectifs de l'État et de l'entreprise dans la société française. J'aurai l'occasion d'y revenir dans les prochaines semaines. Au-delà de ces précisions sur le programme de stabilité, je voudrais aussi redire à quel point toutes les transformations économiques que je viens d'évoquer ne peuvent prendre leur sens que dans une dimension européenne. Innover n'a de sens que si nous rassemblons toutes les capacités d'innovation des grands États européens. Se protéger contre le pillage des technologies par d'autres grandes puissances n'a de sens que si nous le faisons à l'échelon européen. Travailler sur l'intelligence artificielle n'a de sens que si on le fait à l'échelle européenne. Investir dans les supercalculateurs n'a de sens que si l'on y emploie toutes les ressources européennes. Restaurer notre compétitivité sera mille fois plus utile si nous parvenons en même temps à bâtir un marché unique beaucoup plus intégré qui offrira à chacune de nos entreprises, quand elle lancera un produit, non pas 65 millions de consommateurs, mais 450 millions. La profondeur La profondeur de marché que donne l'Europe, c'est de la puissance pour nos entreprises, en particulier pour nos PME ! Faire l'union bancaire, c'est garantir à tous nos concitoyens que l'économie sera stable, que leur épargne sera toujours protégée et qu'ils ne courent aucun risque face aux différentes crises économiques ou financières qui peuvent toujours survenir à un moment ou à un autre. Réaliser la convergence fiscale, achever la zone euro,

nous avançons avec l'Allemagne dans l'intégration de la zone euro. Mon homologue allemand Olaf Scholz et moi-même progressons sur l'union bancaire, sur l'union des marchés de capitaux, sur la convergence fiscale. Nous avançons de la seule manière efficace quand il s'agit du couple franco-allemand

Nous avons tiré la conséquence de ce constat. Nous pensons que l'État doit réaliser plus d'efforts que les collectivités locales, ce qui n'exclut pas que celles-ci poursuivent les leurs.

avec un niveau légèrement inférieur à la moyenne des estimations, mais aussi 2019, l'hypothèse retenue s'établissant ainsi dans la fourchette haute des estimations disponibles. Enfin, sur la période 2020-2022, il est fait l'hypothèse d'une croissance stable. On peut donc considérer que le Gouvernement retient un scénario intermédiaire entre celui du FMI et celui du consensus des économistes

qui devrait vous permettre, si finalement les taux d'intérêt remontaient comme l'anticipent les autres pays, d'absorber d'éventuels dérapages constatés sur les dépenses pilotables

du pacte de stabilité dès cette année, le doute concernant l'exercice 2019 étant en grande partie levé grâce à l'amélioration de la conjoncture. Plus globalement, l'amélioration du contexte macroéconomique devrait permettre un redressement accéléré de la situation des finances publiques au cours du quinquennat. Il convient cependant de s'interroger sur la pérennité de ce redressement, dès lors que le retour à un déficit nominal inférieur à 3 % tient à la reprise économique et

étant insuffisantes pour le contenir. Bien que l'effet des mesures nouvelles en prélèvements obligatoires, hors mesures exceptionnelles, soit neutre en 2017, la part des prélèvements obligatoires dans la richesse nationale

Le présent projet de programme de stabilité maintient toutefois l'objectif initial du Gouvernement de baisse de 1 point de la part des prélèvements obligatoires dans la richesse nationale d'ici à 2022. Avec un taux de prélèvements obligatoires de 44,3 % en 2022, cela resterait malheureusement insuffisant pour revenir sur la hausse observée au cours du précédent quinquennat ; je me tourne, à cet instant, vers le côté gauche de l'hémicycle ... Autre constat, il apparaît que l'amélioration du déficit structurel, qui s'est réduit de 0,5 point l'an dernier, a été essentiellement due aux effets d'élasticités.

validée. Cette règle permet en effet de dépenser jusqu'à la moitié des « bons résultats » constatés en exécution sur le solde structurel. À l'époque, nous avions émis les plus grandes réserves à ce sujet, considérant que, s'il devait y avoir de meilleurs résultats

Parallèlement, l'effort structurel en dépense se révèle négatif, pour la première fois depuis 2012. En outre, l'année 2018 est marquée par un objectif de maîtrise de la dépense moins ambitieux. En effet, lors du débat d'orientation des finances publiques

La nouvelle trajectoire 2018-2022 proposée au travers du présent projet de programme de stabilité doit s'inscrire dans le respect de nos engagements européens, alors que, même si les choses vont mieux, la France se trouve dans une situation atypique par rapport à ses partenaires européens, notamment au regard de son niveau de déficit et de dette publics.

Monsieur le président, messieurs les ministres, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général de la commission des affaires sociales, mes chers collègues,

car il s'agit non pas d'un simple document prévisionnel, mais des engagements européens de notre pays. Je pense d'ailleurs qu'il faudrait lier cet exercice de projection de nos finances publiques à l'arrêté des comptes de l'année passée, toutes administrations publiques confondues, afin de tirer toutes les conséquences de l'exécution budgétaire. Nous en reparlerons sans doute avec le Gouvernement dans le cadre de notre réflexion sur l'amélioration de nos procédures budgétaires. J'en viens au programme de stabilité, désormais quinquennal. La situation économique de notre pays s'améliore, c'est indéniable : l'environnement international est « porteur », la demande intérieure est « dynamique », la progression de l'investissement des entreprises est « historique

les fruits de cette croissance, à la fois pour redresser nos finances publiques et pour financer nos priorités nationales. Les réformes fiscales que vous avez vous-même engagées, la transformation de l'impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière, la création du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital, la disparition progressive de la taxe d'habitation viennent à peine d'entrer en vigueur ou n'interviendront progressivement qu'à compter de l'automne. Ce ne sont donc pas ces réformes qui expliquent notre dynamisme économique au cours de l'année écoulée. L'amélioration économique résulte autant du contexte international et de la reprise dans la zone euro- le taux de croissance, s'établissant à 2,5 %, a atteint son plus haut niveau depuis dix ans -que des mesures prises par le précédent gouvernement, qui ont permis à notre pays de retrouver un chemin de croissance. Ce ne sont pas non plus les mesures budgétaires que vous avez prises depuis six mois, comme la baisse du nombre des contrats aidés ou des subventions au logement social, qui entrent en vigueur cette année, qui peuvent expliquer le redressement de nos finances publiques. Nous ferons plus tard le bilan de ces mesures pour savoir si elles contribuent réellement à augmenter notre potentiel de croissance et nous attendons de voir ce que pourra donner le processus « Action publique 2022 » en termes d'amélioration de l'action publique Vous ne pouvez donc pas revendiquer le mérite exclusif du passage de notre déficit public sous la barre des 3 % du PIB en 2017. Nous nous en réjouissons tous, mais la vérité est que notre déficit, qui atteignait 5 % du PIB en 2012, a été progressivement réduit depuis cinq ans, malgré un contexte économique bien moins porteur qu'aujourd'hui, jusqu'à atteindre déjà 3,4 % à Les mesures en dépenses décidées depuis l'audit alarmiste de la Cour des comptes se sont limitées à 0,2 point de PIB, ce qui correspond à une procédure de régulation classique.

du PIB -, alors même que la baisse de l'impôt sur les sociétés se poursuivrait, de même que la baisse des charges pour les entreprises. Entendez-vous réellement autant alléger la pression fiscale des ménages que celle des entreprises et des patrimoines les plus importants ? trace de la manière dont vous escomptez financer la perte de recettes de 10 milliards à 14 milliards d'euros liée à la suppression progressive de la taxe d'habitation. Par ailleurs, d'autres prélèvements pèseront fortement sur les ménages, y compris les plus modestes, notamment au titre de la CSG et de la montée en charge de la fiscalité écologique. l'OFCE, a démontré que les mesures nouvelles pour les ménages que vous avez fait adopter profiteront largement aux 2 % de ménages les mieux lotis au regard de la distribution des revenus, qui détiennent l'essentiel du capital mobilier. Cette stratégie sera-t-elle poursuivie ? Pouvez-vous nous donner des éléments sur le caractère redistributif de la politique fiscale que vous menez ? Comment comptez-vous mettre en place une réelle évaluation de ses résultats, à l'instar de ce qui a été fait par le passé pour le crédit et l'emploi ? La répartition des efforts en dépense entre les administrations publiques constitue le deuxième sujet. Votre trajectoire implique un fort ralentissement de la dépense locale, par une pression sur la masse salariale, les effectifs et les dépenses de fonctionnement. Il conviendra de voir si la contractualisation qui se met en place le permet, sans entraver la libre administration locale. Votre trajectoire suppose également une progression modérée des dépenses de sécurité sociale. Hormis l'effet de la croissance économique, comment entendez-vous redresser les comptes sociaux dans un contexte de vieillissement de la population et d'accroissement des Pour les années 2019 à 2022, le Haut Conseil des finances publiques considère que le scénario de croissance retenu est optimiste. Nous ne sommes pas à l'abri de nouveaux ralentissements, et des précautions s'imposent. La dette est le troisième et dernier

monsieur le rapporteur Monsieur le président, messieurs les ministres, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général de la commission des finances, mes chers collègues,

Naturellement, je centrerai mon propos sur la trajectoire envisagée des comptes des administrations de sécurité sociale, les ASSO. Le projet de programme de stabilité prévoit une contribution constamment positive des ASSO au solde public sur l'ensemble de la période

On notera cependant que la méthode de calcul actuelle intègre des « bénéfices » qui n'en sont pas vraiment et qui ne permettent quoi qu'il en soit en aucun cas le financement de dépenses courantes. Je pense aux 14,3 milliards

16,3 milliards d'euros, cela correspond précisément à 0,73 point de PIB. Dès lors, on voit bien qu'un tel écrêtement

Ce manque de détail concerne d'abord la distinction entre solde structurel et solde conjoncturel, qui ne se fait pas au niveau des sous-secteurs. Or, d'une part, le Haut Conseil des finances publiques considère que la prévision de croissance du Gouvernement pour 2020-2022 est « optimiste ». D'autre part, « optimiste ». D'autre part, les comptes sociaux sont très sensibles à la conjoncture, en recettes comme en dépenses. Au-delà, on peut se demander à quoi sert d'établir une telle distinction dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques sans possibilité d'en effectuer un suivi sérieux.

entre ces deux périmètres pour la période à venir. Cette lacune nous pose un problème sérieux, puisqu'elle empêche le Parlement, au moment de l'examen du PLFSS, de voir si le projet de loi s'inscrit, ou non, dans la trajectoire que nous avons définie.

Le projet de programme de stabilité reste elliptique sur ce sujet. En tout cas, il ne faudrait pas qu'un « fétichisme » de l'ONDAM se traduise par un transfert de déficit et de dettes vers d'autres acteurs publics, comme les hôpitaux. Nous y veillerons. S'agissant de l'assurance-chômage, comment une norme sévère de dépenses sociales sera-t-elle compatible avec l'ouverture de nouveaux droits pour les personnes qui démissionnent ou pour les indépendants ? Nous n'avons aucune information sur ce point ; cela reste pour nous un mystère. En conclusion, monsieur le ministre, la commission des affaires sociales se réjouit de l'amélioration des comptes publics et vous soutiendra pour poursuivre dans cette voie, mais elle maintiendra sa vigilance, autant que les outils à sa disposition le lui permettront ... À cet égard, puisque « efficacité » semble être devenu le maître mot pour juger de l'action des pouvoirs publics, permettez-moi de vous dire qu'améliorer les outils de pilotage et d'évaluation du budget de la sécurité sociale et des comptes des ASSO serait sans doute bien plus efficace que réduire de vingt jours l`examen du budget au Parlement ou organiser l'examen commun, forcément artificiel,

-objectifs évaluatifs d'un côté, crédits limitatifs de l'autre. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler dans les mois à venir. La parole est

nous serions sur la bonne voie et, grâce au train des réformes, qui traduisent autant d'engagements de campagne, le pays devrait bientôt goûter aux félicités de l'équilibre budgétaire. Vous avez dit « réduction du déficit budgétaire », « réduction des déficits en format européen » mais la réduction du déficit provient autant de la maîtrise des dépenses que de la progression des recettes. J'ai encore souvenir, mais cela n'a évidemment pas été rappelé, que nous avons voté cet automne un collectif budgétaire prévoyant, « brut de décoffrage », 5 milliards d'euros de recettes nouvelles au titre de l'impôt sur les sociétés acquitté par nos plus grands groupes industriels et commerciaux. La chose a certes fait couiner quelques grands groupes économiques, mais on ne saurait oublier que que l'année boursière 2017 s'est achevée sur l'annonce de 94 milliards d'euros de bénéfices cumulés pour les entreprises du CAC 40 : on le voit, du capital, il y en a dépendantes, les EHPAD, les surveillants de prison, les magistrats, les élus locaux, les retraités, les infirmières, bien d'autres encore attendent avec une impatience non dissimulée, ces temps-ci, les effets tant espérés du « ruissellement ». À la vérité, la stabilité ne s'applique guère aux dividendes et aux profits. Malgré la croissance, qui serait retrouvée, et le retour de l'inflation, qui risque de faire sentir ses effets sur les taux longs, sans parler de la guerre économique et fiscale relancée ces derniers temps par M. Trump à Washington, comme est fragile le résultat obtenu ! Les signes ne trompent pas et ils devraient interpeller. Nous conservons un déficit primaire important. déficit primaire important. En clair, cela signifie qu'une fois payés les dépenses de fonctionnement et les intérêts de la dette, nous sommes encore en déficit et que nous n'avons plus d'argent pour investir dans l'avenir du pays.

largement ouvert à la concurrence, laquelle, comme nul ne l'ignore, fait baisser les prix et stimule l'innovation ... L'amélioration du solde budgétaire est donc trompeuse. Elle masque fort mal les restrictions de crédits, comme d'ailleurs les cadeaux fiscaux qui continuent d'être prodigués à ceux qui n'en ont pas besoin et alimentent le robinet du « ruissellement ». La dépense publique, La dépense publique, qui finance l'éducation, les dépenses de santé, la formation, la recherche, contribue elle aussi, qu'on le veuille ou non, à la croissance et au progrès économique. Elle n'est pas nuisible par nature, elle est aussi un levier. Je pourrais également évoquer la situation des comptes des collectivités locales, eux aussi en excédent en raison d'un ralentissement significatif des investissements locaux, mais il est temps, mes chers collègues, que nous parlions enfin d'autre chose.

Nous ne siégeons pas au Parlement pour discuter tous les ans de l'amertume de la purge que les marchés financiers imposent aux populations, des attentes et des aspirations de ceux-ci en vue de garantir au mieux la rentabilité du capital. Il y a des objectifs politiques plus audacieux, mes chers collègues. Il est temps de mettre un terme aux logiques d'arriération des politiques budgétaires actuelles. La question qui se pose avec une acuité forte aujourd'hui, c'est celle de l'indispensable modification de la répartition de la richesse produite dans ce pays.